une soixantaine de duos constitués de nos collègues, de collaborateurs ou de membres du personnel et de personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir le fonctionnement de notre institution et nos métiers. Le Sénat est pleinement mobilisé pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, notamment au travers de ces journées d’échanges, qui constituent un moment privilégié pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés. Je remercie chaque sénateur, sénatrice, fonctionnaire, contractuel et collaborateur de sa participation à cette journée consacrée à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Au nom du bureau du Sénat, j’appelle chacun d’entre vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Fidèle à la Constitution, le Sénat est la maison des collectivités locales, une maison ouverte toute l’année à tous les élus qui maillent nos territoires, avec dévouement et responsabilité, que ce soit en métropole, en outre mer, mais aussi aux conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger,

Sur nos travées, dans cet hémicycle, malgré nos sensibilités différentes, nous savons ensemble défendre les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Monsieur le Premier ministre, vous savez comme nous ce dont tous les élus ont besoin, quel que soit l’échelon auquel ils exercent. Nous y travaillons au Sénat : un statut qui protège la fonction d’élu ; un cadre simplifié pour l’exercice des compétences locales ; une clarification, bien sûr, des règles d’autonomie financière. Assises des départements de France, vous avez indiqué que le modèle départemental est arrivé à ses limites. Peut on aujourd’hui en savoir plus sur votre projet d’instance de pilotage partagée ? Les départements jouent un rôle incontestable de bouclier social. Au fil des crises, ils investissent de plus en plus de moyens pour soutenir nos concitoyens dans la proximité, y compris pour aider nos agriculteurs, qui lancent en ce moment même un nouvel appel de détresse.

à bout. On constate – et c’est le sentiment des conseillers départementaux aujourd’hui – qu’ils se sont transformés en distributeurs de subventions obligatoires,

décidé ensemble, pour plusieurs années. Les départements, comme les communes, ont besoin de prédictibilité et de visibilité. J’ai annoncé un certain nombre de mesures, qui sont en discussion en ce moment même devant votre assemblée, pour améliorer la copie,

évoqué la proximité naturelle entre les départements et le monde agricole et rural, qui souffre et exprime aujourd’hui des incompréhensions, des colères, des demandes. J’ai à mes côtés Annie Genevard, la ministre de l’agriculture, en qui j’ai confiance et qui travaille énormément pour répondre à la colère et aux inquiétudes des agriculteurs.

Chacune de ces surtranspositions, quand elle n’est pas justifiée, introduit de la concurrence déloyale,

et Républicain. Monsieur le Premier ministre, les maires de France, nombreux dans nos tribunes aujourd’hui, devront ils demain augmenter le tarif de la cantine dans leurs écoles ou bien réduire le grammage des repas distribués aux enfants ?

les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron ont détricoté, maille après maille, le contrat constitutionnel entre l’État et nos collectivités. Votre gouvernement, monsieur le Premier ministre,

les élus locaux ne sont pas dupes de vos astuces politiciennes. Ce n’est pas parce que ces coupes budgétaires seront moins élevées qu’annoncé que nous les accepterons. Notre position ne changera pas : baisser les moyens des collectivités, c’est non ; s’attaquer au reste de leur autonomie financière, c’est encore non, pas par corporatisme, mais parce que nous sommes convaincus qu’affaiblir les communes est une faute politique. C’est se priver de leur rôle historique d’amortisseur de crise. C’est se priver de leurs investissements pour l’aménagement du territoire et le bien être de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, nous ne vous laisserons pas fracasser l’avenir des communes sur le mur de votre incurie budgétaire. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple : comptez vous poursuivre cette politique de casse de la décentralisation, au risque de conduire à une crise non pas des « gilets jaunes », mais des « écharpes tricolores »

aucune atteinte à l’autonomie financière des collectivités territoriales ! Monsieur le Premier ministre, votre politique vise à mettre à genoux les élus de la République à l’échelon local : nous serons là pour les maintenir debout

Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles nous avons appelé à cet effort l’ensemble des partenaires, des collectivités et des citoyens, en essayant d’être justes. Je ne suis pas sûr que nous ayons

Union Centriste. Monsieur le ministre de l’intérieur, connaissez vous Rumilly ? Ville de 16 000 habitants située dans le département de la Haute Savoie, aux confins de la Savoie, monsieur le Premier ministre, entre Annecy et Aix les Bains, En plein après midi, et au centre ville, une bagarre générale entre deux bandes rivales s’est soldée par la mort d’un jeune de 17 ans, tué d’une balle dans la tête. Un autre jeune, blessé au thorax, est actuellement entre la vie et la mort. Je pense à leurs familles et je comprends le traumatisme que cela représente pour les habitants de Rumilly et pour les élus de cette ville. L’enquête déterminera bien sûr si cette affaire est un règlement de comptes et/ou si elle est liée à des trafics de stupéfiants. En tout état de cause, ce drame est la preuve que même nos petites villes n’échappent pas aux phénomènes d’hyperviolence. Monsieur le ministre de l’intérieur, les Français aspirent à la paix dans l’espace public. Alors que les maires de France se réunissent pour leur congrès annuel à Paris, quelles sont les initiatives prises par le Gouvernement pour les soutenir dans leurs actions locales visant à préserver la sécurité de nos concitoyens et à prévenir les violences ?

des violences de plus en plus désinhibées, des violences dont les auteurs et les victimes sont de plus en plus jeunes, des violences qui sont en train

Nous ne réglerons pas la question de l’hyperviolence avec des coups de menton ; nous ne la réglerons pas non plus en claquant des doigts. L’État seul ne pourra pas la régler. la régler. Je l’ai dit ici il y a quelques jours en réponse à une question, nous avons réuni l’ensemble des acteurs de l’État chargés de la sécurité publique : les préfets, les policiers, les gendarmes. Je leur ai demandé d’élaborer, sur le terrain, un plan d’action pour restaurer la sécurité publique. C’est un contrat entre eux et nous. Je vais leur donner plus de liberté, en échange de résultats. Je leur ai surtout demandé de travailler avec les élus locaux, dans un continuum de sécurité. C’est fondamental. Je viens de visiter deux communes, Meaux et, en Moselle, Metz. Je vous assure lorsque les élus se sentent concernés, quand ils réunissent, notamment au sein de comités locaux de sécurité, l’ensemble des partenaires, les policiers, bien sûr, les gendarmes, mais aussi la justice

Monsieur le ministre, merci d’aider Rumilly ! Merci d’aider toutes les communes de France face au défi de l’insécurité. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Amateurisme ou insincérité ? Le résultat sera le même : néfaste. Ce gouvernement sera t il celui de l’abandon par l’État des collectivités territoriales et des services au public ? Assumez vous de mettre en péril ces piliers de la République que sont les communes pour laver les péchés d’une politique budgétaire nationale coupable du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

la péréquation, puisqu’elles reçoivent une aide et ne participent pas. En d’autres termes, toutes les communes de France n’étaient pas directement concernées, sauf

L’autre réalité de ce budget est que la majorité sénatoriale est prête à lâcher les collectivités territoriales et les politiques locales qui touchent directement les habitants, et ce sous couvert de responsabilité et sous prétexte de certaines petites avancées que vous appellerez des victoires.

Ce texte comporte des dispositions opérationnelles pour régler les difficultés de nos communes tout en respectant l’effort de sobriété foncière et, bien sûr, la nécessité de prendre des mesures

on sait ce que c’est qu’une trace durable. Et on aime les chemins, même escarpés ! Je ne parle pas du travail du Premier ministre…

monsieur le président, je vous dirai d’emblée, sans ambiguïté, que nous ne renoncerons pas à l’objectif de sobriété foncière. Nous devons maîtriser les risques d’une excessive artificialisation des sols. sols. Je n’ai pas oublié les catastrophes auxquelles nous avons dû faire face. Il y en a eu un certain nombre au cours des dernières années. Je ne parle pas seulement de ce qui s’est passé à Valence, dans un pays voisin et ami. N’ayons pas la mémoire courte,

En même temps, on constate que la législation, la réglementation, enserre les maires dans un carcan. Or ceux ci doivent pouvoir exercer leur mission, qui est aussi d’être des maires bâtisseurs,

mais nous devons aussi construire le ZAN en partant davantage de la réalité des besoins et du dialogue avec chaque territoire. En attendant, nous allons prendre, sous l’impulsion de Catherine Vautrin, plusieurs dispositions pour apporter de la souplesse, avant même le vote de ce texte, là où c’est possible et nécessaire. Nous inviterons les préfets à se saisir de la circulaire dite des 20 %, afin de donner des marges supplémentaires aux collectivités territoriales qui en ont besoin immédiatement. plus, nous allons modifier les décrets pour que les jardins pavillonnaires ne soient plus considérés comme des surfaces artificialisées. Nous prendrons aussi en compte les nouveaux projets au titre des projets d’envergure nationale et européenne. Je veillerai à ce que les préfets soient informés de notre volonté de changer bientôt la loi

mais aussi faire attention à l’environnement. La

La parole est à M. Saïd Omar Oili, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre

estiment entre 6 000 à 10 000 le nombre d’enfants non scolarisés, soit 9 % du total. Les chiffres que je viens de vous citer émanent de la chambre régionale des comptes de Mayotte et des services de votre ministère. Ces données illustrent très bien l’origine de la progression, fulgurante ces dernières années, de la délinquance juvénile. on peut s’interroger sur le lien entre cet état des lieux et le caillassage des bus scolaires, les intrusions et les tentatives d’incendie des établissements scolaires, qui sont le quotidien des habitants de Mayotte. Hier matin encore,

le ministère de l’éducation nationale compte t il prendre face à cette situation aux conséquences d’ores et déjà catastrophiques pour l’avenir de Mayotte et de ses générations

le gouvernement de M. Barnier, notre Premier ministre, seront à vos côtés pour soutenir Mayotte, parce que l’école est notre priorité nationale. Nous devons à tout prix élever le niveau de tous et ne laisser personne sur le bord de la route, sans excepter nos jeunes Mahorais. Soyez assurés de notre complet soutien. Nous serons à vos côtés tout au long de l’année 2025 et des années qui viennent pour que le territoire de Mayotte et nos jeunes Mahorais fassent partie de la promesse républicaine, de la promesse d’avenir de la Nation. La parole est à Mme Laure Darcos, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Il faut dire que leur confiance envers l’État a maintes fois été érodée par la question des compensations à l’euro près, l’inflation normative ou encore la diminution considérable de leur autonomie financière. Alors que nos collectivités territoriales ont l’obligation de présenter des budgets équilibrés en recettes et en dépenses, elles ont été désignées l’été dernier parmi les responsables des déficits publics catastrophiques de notre pays.

Or n’oublions pas que nos élus sont les premiers investisseurs publics, qu’ils portent à bout de bras la modernisation de nos infrastructures locales, dédiées à nos populations et à notre économie, et qu’ils font face aux enjeux majeurs de la parentalité ou de la transition écologique. Pouvez vous nous assurer que les sommes qui seront prélevées à une collectivité territoriale lui seront bien restituées intégralement au 1 janvier 2026, et qu’il ne s’agit pas d’un fonds de péréquation déguisée ? Par ailleurs, pouvez vous nous confirmer que ce mécanisme ne sera pas étendu à d’autres collectivités dans le cas où les finances publiques se dégraderaient encore ? Certes, il est nécessaire que chacun contribue aux efforts pour assainir les finances publiques, mais ces efforts doivent être justement répartis et ils ne doivent pas pénaliser les plus vertueux. La parole

Chaque année, ils sont environ 450 à jeter ainsi l’éponge, usés par les menaces, les insultes, les attaques physiques, le climat étouffant créé par des individus agressifs. Dans la Creuse, un homme a été condamné en juin dernier après avoir déclaré au maire de sa commune : « Une mairie, ça brûle bien ! » Le mois dernier, un député a reçu des injures puis des coups de poing dans le ventre à la sortie d’un supermarché où il faisait des courses avec sa fille. Une telle bestialisation ne peut que nous plonger dans la consternation. Une étude parue vendredi dernier dresse un portrait très alarmant de la santé mentale des maires : 83 % d’entre eux estiment que leur mandat est usant pour leur santé, et près de la moitié songe fréquemment à démissionner. L’ampleur et la gravité de ces faits appellent une réponse volontaire du législateur pour sauvegarder le fonctionnement ordinaire de la démocratie locale. Au cours d’un échange que vous avez eu récemment avec le président Mathieu Darnaud, vous avez évoqué votre intention d’adresser une nouvelle circulaire aux procureurs généraux et aux procureurs de la République afin de mettre à leur disposition de nouveaux outils pour lutter contre ces violences. Le plan national de prévention et la loi du 21 mars dernier ont renforcé l’information des maires sur les infractions et ont consolidé le dialogue entre parquets et collectivités Pourtant, le résultat n’est pas encore à la hauteur de nos attentes. Ma question est la suivante : quelles sont vos pistes pour assurer, une bonne fois pour toutes, la sécurité de nos élus ?

Attaquer des élus, c’est attaquer la République. Cela n’est pas supportable, et cela appelle de la part de l’État et de la justice une réponse extrêmement ferme.

Vous le savez, la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a permis d’élargir le spectre des atteintes aux élus en incluant de façon pertinente, les candidats, en allongeant certaines durées de peine ou en parachevant les mécanismes juridiques d’information des élus.

Nous avons adressé aux procureurs généraux un modèle de protocole relatif au renforcement des relations entre les parquets et les maires. Je souhaite évaluer l’efficacité de l’ensemble des mesures que nous avons prises.

les parlementaires. En tout cas, soyez assuré de ma pleine mobilisation et de la pleine mobilisation de la justice pour que les menaces contre les élus puissent être poursuivies et sanctionnées avec la plus grande fermeté.

et Républicain. Monsieur le Premier ministre, c’est la double peine pour les communes, pour les employeurs territoriaux et hospitaliers. Lors des Assises des départements de France, vous avez affirmé vouloir redonner des marges de manœuvre, de l’oxygène, de la liberté aux collectivités territoriales, afin de restaurer le sens de leur mission.

Au lieu de restaurer leurs missions, vous les contraignez à réduire leurs services essentiels sous le poids d’une pression financière insoutenable. Toutes les communes seront touchées. Toutes les collectivités territoriales seront concernés. Comment justifiez vous cette contradiction ? Comment pouvez vous parler de redonner de la liberté aux collectivités territoriales tout en les étranglant financièrement, sans même leur offrir la moindre concertation sur le sujet ? Vous le savez, c’est là une décision unilatérale du Gouvernement.

Avec ces nouvelles charges de fonctionnement, l’autofinancement se réduit comme peau de chagrin. Il est grand temps de passer des mots aux actes et de rétablir un véritable dialogue avec les collectivités locales, avant qu’il ne soit trop tard.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour le groupe Les Républicains.

C’est le quotidien des Françaises et des Français. Je le rappelle, les dépenses des collectivités ne représentent que 19 % de la dépense publique totale, contre 34 % en Europe, alors que celles ci assument 70 % de l’investissement public, pour seulement 8 % de la dette. Même si chacun doit contribuer en responsabilité à un effort consenti pour redresser nos comptes publics, nous attendons de l’État que cet effort soit juste et soutenable. La priorité doit donc être de garantir l’épargne des collectivités, qui produit immédiatement un investissement dont notre pays a besoin.

Ensuite, supprimer toute mesure rétroactive et garantir lisibilité et stabilité des relations avec les collectivités ; je pense évidemment d’abord au FCTVA. Enfin, et peut être surtout, renoncer à capter l’épargne des collectivités tout en la gelant pour partie dans leurs comptes ; je pense en l’occurrence aux modalités du fonds de précaution, qu’il faut profondément modifier en faisant confiance aux collectivités. Monsieur le ministre chargé du budget, vos réponses pourront se traduire en amendements dès la semaine prochaine, et ainsi éviter un blackout territorial et amorcer le contrat de confiance, tel que le Premier ministre le souhaite et nous y invite. La

Monsieur le ministre, notre sécurité civile repose sur un modèle qui démontre chaque jour sa pertinence et son efficacité, en associant les sapeurs pompiers professionnels et les sapeurs pompiers volontaires au service d’un même objectif : protéger la population, les biens et l’environnement. Par son organisation, notre modèle de sécurité civile nous permet de faire face aux accidents du quotidien comme aux situations de crise exceptionnelles. Nous l’avons malheureusement encore constaté voilà quelques semaines, notamment dans le département de la Haute Loire.

de retraite au titre de la solidarité nationale pour reconnaître leur engagement citoyen et favoriser leur fidélisation. Vingt mois après l’adoption du texte, cette mesure, votée à l’unanimité sur nos travées, n’est toujours pas effective, faute de décret d’application. Le 13 décembre dernier – cela fait pratiquement un an –, votre prédécesseur, répondant à une question de mon collègue Pascal Martin, indiquait sa volonté d’avancer sur le sujet. de septembre, lors du congrès des sapeurs pompiers de France, à Mâcon, M. le Premier ministre a rappelé la volonté du Gouvernement de mener à son terme ce travail interministériel. Monsieur le ministre, quand pourrons nous exprimer à nos sapeurs pompiers la reconnaissance qui leur est due au titre de leur engagement ?

La parole est à M. Christian Bruyen, pour le groupe Les Républicains.

Je prends cet exemple non pas pour déplacer le problème, mais afin d’organiser la répartition des vols et, ainsi, de ne pas dépasser le seuil d’acceptabilité des populations concernées. Les opérateurs terrestres ne s’en plaindront pas, tant certains se sentent « maltraités », en termes d’immobilisation au sol du fait de l’engorgement des plateformes franciliennes. En outre, est il acceptable que du fret français soit traité à l’étranger

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces éléments de réponse, qui me donnent un peu d’espoir. Manifestement, le sujet vous préoccupe. Les perspectives d’évolution se font jour. Il convient d’aller plus loin, avec des solutions pérennes. Ce n’est pas facile, j’en conviens, mais nos voisins travaillent de façon très prometteuse. Je pense à Amsterdam, avec Maastricht, à Bruxelles et à d’autres. La France doit faire de même. La souveraineté économique tient aussi à la maîtrise des approvisionnements

La parole est à Mme Marion Canalès, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. et Républicain. Les réseaux sociaux sont devenus le nouvel eldorado des atteintes à l’intégrité des individus, et les élus ne sont pas épargnés. Un maire sur quatre en a été victime. Si l’intelligence peut être artificielle, la violence qu’elle induit est, elle, bien réelle. Un clic peut blesser plus qu’un coup. Voilà quatre jours, le visage d’un député du Puy de Dôme a été découpé en deux au couteau, tandis que la tête du maire de Clermont Ferrand et celle d’un adjoint étaient écrabouillées dans une presse. À celles et à ceux pour qui ces montages ne seraient « pas si dramatiques », nous devons répondre fermement que l’intelligence artificielle générative crée des contenus toujours plus extrêmes, augmentant le risque de passage à l’acte. Nous ne devons pas banaliser l’intolérable, même en ligne ; les plaintes doivent être suivies d’effets. Dans 500 jours auront lieu les

plus d’interlocuteurs. C’est donc aux maires qu’ils s’adressent : le « dernier à portée d’engueulades », comme ils disent. Chaque décision gouvernementale qui affaiblit la capacité de faire des élus locaux est un coup de canif supplémentaire porté dans le contrat passé avec eux et la République. Affaiblis, plus vulnérables, les élus locaux se sentent plus démunis. Dépourvus de moyens, ils deviennent, aux yeux de leurs détracteurs, de mauvais gestionnaires, voire inutiles, et ils ne mériteraient plus que du mépris.

Je me réjouis que ce gouvernement s’occupe enfin du sujet très préoccupant de la surexposition des enfants aux écrans, notamment des tout petits. C’est un sujet sur lequel, forte d’un rapport réalisé au nom de notre la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport en 2018, j’avais alerté votre prédécesseure Agnès Buzyn.

laissait penser qu’il s’agissait d’une urgence nationale. Aujourd’hui, les études le démontrent, le phénomène tend à s’aggraver : retards dans l’apprentissage ; difficultés d’attention et de concentration ; attitude passive de l’enfant face au monde qui l’entoure. Au delà des mesures sectorielles que vous avez annoncées, quel plan global de prévention et d’action, associant élus, professionnels de santé, familles, enseignants et éducateurs, et en prenant appui sur l’ensemble de nos propositions, entendez vous mener avec vos collègues membres du Gouvernement chargés de l’éducation nationale, de la petite enfance et du numérique ?

La séance est reprise. La parole est à M. Bernard Jomier, pour un rappel au règlement.

Il nous paraîtrait utile, notamment sur le premier sujet, et alors que nous n’avons pas fini de discuter des exonérations de cotisations sociales, que les termes du débat soient stabilisés, de sorte que nous puissions nous prononcer en connaissance de cause. Nous avons volontiers salué la volonté manifestée par le Premier ministre, après des

en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités et la gestion des risques économiques, patrimoniaux, fiscaux, écologiques et sanitaires associés. En application de l’article 8 , alinéa 5, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Cet amendement tend à placer les entreprises ultramarines du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) dans un barème renforcé d’exonération de charges pour deux années, en raison des difficultés majeures qui fragilisent ce secteur dans nos territoires. La filière réunionnaise du BTP, par exemple, a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en dix ans. Cet allégement temporaire constituerait un signal fort pour soutenir l’activité et préserver l’emploi dans un secteur essentiel pour les économies locales. La parole

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours, en sus de celles qui sont prévues par le plan d’étalement de la dette. La parole est à Mme Annick Petrus,

Ce mécanisme suspendrait les majorations et pénalités de retard pour les employeurs respectant les échéances. Il s’inspire des dispositifs appliqués après les crises Irma et covid 19.

rétroactivement. Pour les entreprises du BTP, particulièrement affectées par les retards de paiement des collectivités, le remboursement des dettes pourrait être reporté jusqu’au déblocage des fonds publics, sous réserve de justificatifs.

les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés – au delà de 1,6 Smic – n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité

Des travaux ont été menés en lien avec la profession agricole et la Mutualité sociale agricole (MSA), afin d’identifier des solutions pour résoudre les problèmes d’ordre technique, juridique, informatif, liés à la mise en place de cette assiette contemporaine.

On sait tous quels sont les niveaux de rémunération des apprentis. Cette mesure leur ferait perdre entre 50 euros et 100 euros, soit 10 % de leur rémunération.

n’évoquerai pas, car ce n’est pas le sujet aujourd’hui, la casse des lycées professionnels, qui conduit à développer considérablement l’apprentissage. En conclusion, si nous sommes favorables à une réduction de la voilure, pour les raisons que j’ai invoquées, sur les exonérations

Mizzon, sur l’article. Je prends la parole à ce stade pour dénoncer non pas une injustice, mais une inégalité de traitement injuste

par nos collègues. Sans surprise, puisque cet article est le pendant de l’article 6, dont nous avons défendu hier soir la suppression. L’article 7 revient en effet sur plusieurs mesures de soutien à l’emploi, notamment des plus jeunes, en prévoyant d’assujettir à la CSG CRDS

avec près de 850 000 nouveaux contrats enregistrés sur l’année. Je rappelle quand même qu’ils étaient 350 000 en 2017. Cet article 7, qui va de pair avec la baisse des aides versées aux entreprises, dont nous aurons à débattre lors de l’examen du projet de loi de finances, nous semble aller à contre courant des politiques menées en faveur de l’emploi et de l’insertion des jeunes. Le signal envoyé est donc désastreux. Il en va de même pour les jeunes entreprises innovantes. Toute mesure d’économie sur ce dispositif pénaliserait les start up et PME innovantes, alors que l’écosystème subit une crise de financement depuis bientôt deux ans. Cette mesure d’économie interviendrait par ailleurs quelques mois seulement après l’extension du dispositif aux jeunes entreprises de croissance.

une expression consacrée initialement à la Constitution. J’ai été directeur général d’une grande chambre de métiers, la chambre de métiers d’Alsace, au temps béni où l’Alsace était encore une région, et je voudrais toute l’importance que peut avoir l’apprentissage, non seulement en matière d’insertion professionnelle, mais aussi en matière de qualification professionnelle, ce dont parlaient les orateurs précédents. En Alsace, nous avions cette chance, de par notre histoire, d’avoir

pour eux, souvent discriminés qu’ils étaient à leur entrée dans le monde professionnel. La proposition gouvernementale d’élargir le nombre d’apprentis assujettis aux cotisations sociales est une erreur manifeste. Vous connaissez notre position sur les exonérations. Elles ne doivent être conservées que lorsqu’elles sont efficaces. Or réduire les revenus des apprentis dès que leur rémunération dépasse la moitié du Smic, soit moins de 700 euros net mensuels, c’est à dire presque le RSA, attaque directement leurs moyens de subsistance. Il est complètement injuste de faire porter les dérives budgétaires les apprentis, dont nous connaissons la précarité des conditions de vie. Par ailleurs, cette mesure aura un impact important sur la capacité des artisans et petits commerces d’engager des apprentis, car les TPE et PME n’ont pas toutes les moyens d’augmenter la rémunération brute de leurs apprentis pour conserver leur attractivité vis à vis des jeunes. Beaucoup ont proposé, en découvrant cet article 7 dans le PLFSS, de limiter cette mesure aux apprentis de niveau bac ou d’un niveau inférieur à bac+3. Toutefois, il faut garder en tête que deux tiers des apprentis s’engagent dans des études grâce à l’apprentissage, qui est une source de financement des parcours d’études, de plus en plus onéreux. Nous voterons donc la suppression de cet article.

les apprentis ont des droits sans cotiser, alors que les stagiaires paient la CSG CRDS. Or personne ne remet cela en cause.

les dispositions du texte réduiraient le montant de l’aide unique à l’embauche de l’apprenti de 6 000 à 4 500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’État sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, elles, n’ont pas l’obligation d’embauche d’un apprenti.

positifs. En effet, nous avons compté en sept ans plus de 550 000 apprentis supplémentaires, pour atteindre quasiment le million. Pour autant, il me semble que le Gouvernement pourrait modifier quelque peu sa position durant nos débats,

l’amendement n° 283. Les sénateurs RN s’opposent également aux dispositions de l’article 7 du PLFSS 2025, qui visent à réduire les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d’apprentissage, ce qui reviendrait à augmenter le coût d’embauche des apprentis pour les employeurs. Cette mesure risque de compromettre une politique d’insertion professionnelle essentielle pour les jeunes et de freiner la dynamique positive de l’apprentissage. L’apprentissage n’est pas un emploi comme les autres : il s’agit avant tout d’une formation visant à doter les étudiants des compétences nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle future. Sa finalité première est pédagogique ; ce n’est pas la création immédiate de richesses pour l’employeur. Plutôt que de réduire les exonérations sociales, il serait plus judicieux de rationaliser les primes à l’embauche dans le cadre du PLF. Cette approche permettrait de maintenir les incitations essentielles à la formation et à l’insertion des jeunes tout en optimisant les fonds publics pour éviter les véritables effets d’aubaine. Une gestion budgétaire cohérente et réfléchie doit préserver les dispositifs qui soutiennent l’emploi durable et la compétitivité de notre économie. Pour toutes ces raisons, nous demandons également la suppression de l’article 7 du PLFSS 2025. Cette disposition met en péril une politique d’apprentissage qui a démontré son efficacité et sa valeur ajoutée pour l’économie française. La parole

L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qu’il ne faut pas fragiliser, notamment pour nos TPE. Le coût d’apprentissage pourrait augmenter de près de 30 % pour une TPE du bâtiment employant un jeune en CAP si l’article 7 venait à à entrer en vigueur. Cet article arrive dans un contexte déjà particulièrement tendu pour l’apprentissage, le soutien de l’État diminuant fortement avec la baisse des financements de France Compétences. En Lot et Garonne, par exemple, du BTP prévoyait déjà un impact financier de 300 000 euros pour l’année 2025, alors même que la filière accuse une décroissance de 5 % de l’activité. Perte de pouvoir d’achat pour les apprentis, baisse de l’aide unique à l’embauche pour les employeurs : tout le monde est lésé par les mesures contenues dans cet article. Cet amendement vise donc à préserver le système actuel, qui est profitable aussi bien aux jeunes alternants qu’aux entreprises.

Madame Poncet Monge,

partage pas ce point de vue.

Le scrutin est clos.

On vient ici frapper au portefeuille des jeunes engagés dans une démarche de formation et d’insertion. C’est une mesure que je ne peux comprendre au regard du volontarisme des jeunes et des besoins en main d’œuvre de nos artisans. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cette mesure foncièrement injuste pour nos jeunes. La parole

Grâce aux mécanismes d’incitation mis en place par la puissance publique, les entreprises se sont emparées du dispositif, auquel les jeunes ont porté un très vif intérêt. C’est particulièrement le cas pour les TPE et les PME, qui ont ainsi trouvé un moyen efficace de recruter et de former des jeunes. Dans une logique de rationalisation des dépenses publiques, le Gouvernement a fait le choix de restreindre les mécanismes de soutien à l’apprentissage, notamment en assujettissant les rémunérations des apprentis à la CSG CRDS. La hausse du coût du travail des apprentis pourra potentiellement être absorbée par les grandes entreprises, mais elle risque de se révéler beaucoup plus dommageable pour les TPE et les

engagés par des entreprises de plus de 250 salariés.

Les secteurs les plus touchés par les difficultés de recrutement sont le bâtiment et les travaux publics, la restauration et les soins à la personne. Une stratégie de soutien aux apprentis

de CFA deux apprentis ayant la même activité dans deux entreprises différentes ne se voient pas prélever la même part de CSG sur leur rémunération ? Là encore, ce serait une injustice

très différents ! Madame la ministre, soit je me suis mal exprimée, soit vous mélangez deux choses : j’ai indiqué que 8 % des inscrits à France Travail étaient

également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français. Le rapport d’information sur la mise en application de la loi pour l’économie bleue, rendu public au mois de décembre 2017, fait état de l’impact positif de l’élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois

est à Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à maintenir l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur les secteurs concurrentiels des énergies marines renouvelables et des câbles sous marins.

Le dispositif Jeune entreprise innovante (JEI) accompagne la création et la croissance de milliers de PME innovantes sur tous nos territoires. La suppression de la partie sociale de ce dispositif serait délétère pour l’emploi et freinerait la capacité d’innovation française. Elle nous priverait également de solutions pour la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays. Cet amendement vise donc à revenir sur cette suppression et à rétablir le dispositif JEI dans son intégralité, celui ci constituant une part importante de l’architecture de soutien

en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est à dire un impact positif sur les dépenses et sur l’emploi. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse

ne paraît pas souhaitable, car ces exonérations visent à protéger les seules entreprises soumises à la concurrence internationale, c’est à dire celles dont les employés sont les moins qualifiés. Sur les navires de fret hors passagers sur les navires de service, les salaires sont compris entre 2,5 et 4 Smic – et je ne parle pas des entreprises de transport fluvial, dont l’exposition à la concurrence internationale est plus que limitée.

Monsieur le ministre,

Les crédits seraient ouverts en loi de finances pour 2025 à hauteur de ces prévisions : l’impact sur l’équilibre financier de la sécurité sociale serait donc nul. La parole est à Mme

Par cet amendement, nous proposons d’augmenter de 2 points le taux de CSG assise sur le capital. Il s’agit de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche autonomie de la

le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles. En effet, l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 point en 2024 mise à part, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu. Cette réaffectation ne représentera que 2,6 milliards

au financement des caisses de retraite. Depuis plus de dix ans, ces plateformes ont vendu aux travailleurs l’illusion de la liberté et de l’autonomie, alors qu’elles ont en réalité imposé un modèle d’autoentrepreneuriat précaire permettant de s’affranchir des cotisations sociales.

cette situation. S’ils étaient requalifiés en salariés et rémunérés au moins au niveau du Smic, ils pourraient contribuer à hauteur de 1,5 milliard d’euros par an à notre système de solidarité. ces travailleurs ne sont pas indépendants. Ils subissent une subordination économique et algorithmique reconnue par de nombreuses jurisprudences. Aussi, il est urgent d’instaurer une présomption légale de salariat ; nous avons déjà eu

Merci